Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je vous rappelle que l'auteur de la demande du débat dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente. À l'issue

et, d'autre part, d'un nombre croissant d'entrepreneurs qui veulent embaucher, mais qui, faute de trouver les compétences, voire même des candidats, renoncent à des marchés ou à défaut sont contraints à recourir au travail détaché. En 2018, l'enquête besoins en main-d'oeuvre, ou BMO, de Pôle emploi, montre que la pénurie de candidats dans 83 % des cas est le premier motif des difficultés de recrutement, devant l'inadéquation des candidatures et la nature du poste proposé. Ce sont ainsi entre 250 000 à 330 000 offres d'emploi qui n'avaient pas été pourvues

Plus la dynamique de création d'emplois est forte, plus le désajustement entre l'offre et la demande, entre les compétences disponibles et les compétences recherchées, apparaît. Il convient toutefois de rappeler que, dans un contexte d'accroissement fort des offres d'emploi déposées- plus 9,2 % entre la mi-2017 et la mi-2018, soit 3,5 millions d'offres déposées -, une large majorité des offres- plus de 90 % -sont pourvues.

D'autre part, on trouve des métiers où les besoins de recrutement de la part des entreprises sont importants et coexistent avec un nombre significatif de chômeurs, souvent peu qualifiés et avec une forte rotation de la main-d'oeuvre : ouvriers du bâtiment, aides à domicile, serveurs.

la connaissance des métiers, l'incitation au travail, la reconnaissance des métiers et la formation massive pour tirer vers le haut l'ensemble des compétences. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés avec votre concours.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, chaque année, des centaines de milliers d'offres d'emploi ne trouvent pas preneur. À l'heure où le taux de chômage en France est de 9,3 % alors qu'il n'est que de 2,3 % en République tchèque et de 3,4 % en Allemagne et en Pologne, nous pouvons légitiment nous interroger, d'autant que le taux de chômage a baissé dans tous les États membres pour atteindre 6,6 % en moyenne dans la zone euro alors qu'il stagne en France. Nous avons tous en mémoire une phrase qui a fait le buzz « traverser la rue pour trouver du travail ». Derrière cette phrase devenue célèbre se cache une réalité à nuancer. En 2017, Pôle emploi a publié une étude sur les fameux emplois non pourvus. Ces offres restées sans réponse ne le sont pas forcément faute de « gens prêts à travailler ». Sur les 300 000 97 000 d'entre elles ont été annulées par les recruteurs eux-mêmes et 53 000 concernaient des offres toujours en cours. Et si 150 000 recrutements restants ont été abandonnés faute de candidat, surtout faute de profils adéquats, selon cette étude 19 500 offres d'emploi n'ont fait l'objet d'aucune candidature. Enfin, quand on sait que les employeurs ont transmis en 2017 près de 24 millions de déclarations d'embauche, le nombre d'emplois non pourvus prend à cet égard une importance relative. Néanmoins, cette absence de candidatures pose la question de l'inadéquation entre l'offre et la demande. Il existe des secteurs qui peinent à recruter et qui en souffrent. Les candidatures sont inadaptées, les entreprises déplorent le manque de compétences, de connaissances techniques, d'expérience professionnelle ou l'absence d'un diplôme en lien avec le métier. Les principaux postes non pourvus sont ceux d'employés et d'agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration, de cuisiniers, d'assistantes maternelles, de conducteurs de véhicule, de cadres, de technico-commerciaux, d'ingénieurs, de techniciens de l'informatique et de carrossiers. Cette liste ne présente aucune surprise, ces métiers connaissant régulièrement des problèmes de recrutement. Si certains secteurs en tension demeurent, c'est sur eux qu'il faut donc concentrer nos efforts. Ce sont souvent des emplois ressentis comme peu valorisants et/ou peu rémunérateurs, mais aussi des métiers que l'on ne connaît pas vraiment ou qui ont mauvaise presse, comme celui de chaudronnier qui a aujourd'hui peu à voir avec l'image que l'on s'en fait communément. Mon département, la Loire-Atlantique, malgré un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale, ne déroge pas à cette situation. Selon le recensement de Pôle emploi des besoins en main-d'oeuvre pour 2018, plus de 50 % des 54 236 projets de recrutement sont réputés difficiles. Pour 442 d'entre eux, la difficulté est même estimée à 100 %. Dans ces projets de recrutement très difficiles qui représentent donc moins de 1 % du volume global, on retrouve principalement les métiers de charpentier, de régleur, d'ouvrier qualifié industriel, d'ouvrier non qualifié en artisanat, de vendeur en gros, de personnel navigant de l'aviation, d'agent de maîtrise en entretien, de conducteur d'engins, de contrôleur de transports ou encore de concierge. de concierge. Si certaines offres d'emploi ne trouvent pas preneur, c'est peut-être aussi parce qu'elles ne sont pas assez attractives, que ce soit au niveau des missions, du salaire ou au regard de la pénibilité. Quand on recherche un emploi, on privilégie celui qui correspond à son souhait et à sa formation, ce qui est assez légitime. Généralement, le fait d'élargir ses recherches à d'autres secteurs d'activité fait que les niveaux de qualification et de rémunération sont alors moindres. Il est alors difficile pour la personne en recherche d'emploi de se projeter dans un nouveau projet professionnel quand celui-ci, en plus de l'éloigner de son profil initial, est financièrement non stimulant. Enfin, l'attractivité d'un poste dépend aussi des conditions de vie et de la qualité de vie environnante. Entre 2007 et 2011, environ 500 000 personnes ont dû renoncer à un poste en raison de problèmes de logement et du surcoût de la mobilité exigée. exigée. À ce niveau, le mouvement des « gilets jaunes » a mis en évidence dans nos campagnes la problématique du coût de l'essence. Un postulant qui se rend compte qu'aucun logement ne lui sera accessible au regard de ses revenus

C'est un élément très important à prendre en compte, surtout pour les secteurs qui fonctionnent essentiellement en temps partiel et en CDD. La restauration est, de ce point de vue, un bon exemple. Cet environnement favorable est du ressort des collectivités locales, qui doivent penser leur aménagement en ce sens. du ressort des entreprises, qui doivent adapter ces offres non pourvues, notamment en termes de temps de travail, de rémunérations, de mobilité géographique, pour mieux répondre aux possibilités des candidats.

la politique de formation est un enjeu stratégique. La formation professionnelle, initiale et continue demeure donc un enjeu clé. Il est essentiel de mieux cibler les formations et surtout de mieux les adapter aux demandeurs d'emploi. Pour conclure, le chômage n'est pas simplement un choix personnel qui se résoudrait en traversant la rue. Concernant les emplois non pourvus, il ne faut pas se concentrer sur une vaine bataille de chiffres. Le marché du travail est en perpétuelle évolution et a besoin de souplesse. La question fondamentale de la politique de l'emploi demeure l'accroissement du nombre d'offres, pas leur pourvoi intégral ! Néanmoins, pour changer la donne, chacun doit prendre ses responsabilités à l'État de mieux adapter l'offre de formation aux besoins ; aux entreprises de rendre certains métiers boudés par les candidats plus attractifs en termes de salaire, d'horaires ou de conditions de travail ; aux collectivités de faciliter la mobilité géographique liée aux coûts du logement ou des transports.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, alors que le Président de la République a annoncé regretter ses propos blessants à l'égard des Français, nous avons encore toutes et tous en tête la réponse faite à un jeune en recherche d'emploi qui l'avait interpellé sur la question du chômage et auquel il avait répondu : « Je traverse la rue et je vous trouve un emploi »

Pourtant les chiffres sont têtus. Selon Pôle emploi, en 2017, plus de neuf offres d'emploi sur dix ont été pourvues et les offres d'emploi qui n'ont fait l'objet

Nous sommes donc bien loin du compte ! Face à ce « problème », le Premier ministre a déclaré vouloir faire du développement de la formation et de l'apprentissage « une voie royale pour trouver un métier Pourtant, à la demande du Gouvernement, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA, projette de fermer trente-huit centres de formation et de supprimer 1 541 postes en CDI. Avez-vous l'intention, madame la ministre, de laisser fermer des sites

l'AFPA survit chaque année grâce à une aide d'urgence de l'État qui lui permet de boucler son budget. Depuis cinq ans, ce sont plus de 700 millions d'euros de déficit qui ont été accumulés. désespérante à la fois pour les territoires et pour les salariés de l'AFPA, qui ne voient pas l'avenir. La Direction générale de l'AFPA a proposé une réforme structurelle qui va permettre de recentrer cette agence sur des missions plutôt régaliennes

Féret. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour échanger sur un sujet qui fait trop souvent l'objet de questionnements, d'interrogations, voire d'incompréhensions : celui des emplois non pourvus. Pourtant, on le sait, il ne suffit pas de « traverser la rue » et de postuler à un emploi pour être embauché. S'il existe dans certains secteurs, comme ceux du bâtiment, de l'industrie hôtelière ou des services à la personne, un fossé entre demandeurs d'emploi et recruteurs, il n'est pas forcément et exclusivement le fait des premiers. De même, si la plupart des offres d'emploi non pourvues dans ces secteurs le sont en raison de leur manque d'attractivité, la question de la formation- vous l'avez dit, madame la ministre -reste posée. Après le plan de formation de 500 000 chômeurs mis en place par le précédent gouvernement, gouvernement, vous avez lancé le Plan d'investissement dans les compétences, le PIC, avec pour ambition de former 1 million de demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés et 1 million de jeunes éloignés du marché du travail. Nous ne pouvons que saluer cette volonté. volonté. Au regard du projet de loi de finances pour 2019, marqué par la forte contraction des crédits de la mission « Travail et Emploi » pour la deuxième année consécutive, de près de 3 milliards d'euros, et par un affaiblissement historique des différents opérateurs publics chargés de l'accompagnement vers l'emploi, permettez-moi de formuler mes plus vives inquiétudes. Je m'interroge tout particulièrement sur les capacités de ces acteurs à porter le PIC. Prenons l'exemple de Pôle emploi, particulièrement touché, avec une baisse de la subvention pour charges de service public de 85 millions d'euros et l'annonce de la suppression d'au moins 800 équivalents temps plein l'an prochain. Je n'ai pas le temps, malheureusement, d'évoquer la situation des missions locales et des Maisons de l'emploi, elles aussi fragilisées, ni même de revenir sur les difficultés, précédemment évoquées, de l'AFPA, qui montrent bien que la question de l'accompagnement et de la formation des chômeurs dans nos territoires reste posée.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au troisième trimestre de 2018, ce sont 5,6 millions de personnes qui étaient inscrites à Pôle emploi en catégorie A, B et C, parmi lesquelles 3,4 millions étaient sans emploi. Selon une étude de Pôle emploi sur l'année 2017, 300 000 offres n'ont pas été pourvues et 150 000 ont réellement conduit à un abandon de recrutement, faute de candidats. Ces chiffres apportent

Nous constatons également qu'il existe très peu d'emplois non pourvus dans les grandes entreprises, alors que les entreprises de moins de 50 salariés, et de moins de 10 salariés, peinent à recruter. Cela s'explique par le manque de culture « ressources humaines » des TPE. Madame la ministre, nous avons travaillé cet été avec vous sur la formation et l'apprentissage. C'était indispensable. Si nous voulons que ces offres d'emploi trouvent preneur, il convient de rendre ces métiers plus attractifs. Or l'attractivité de ces secteurs n'étant pas constituée du simple fait de l'existence de postes disponibles, il est important de trouver d'autres leviers. Les employeurs expliquent à Pôle Emploi l'insuffisance de recrutement par un manque d'expérience, de motivation ou de compétence des candidats. Une enquête auprès de 5 000 professionnels de l'hôtellerie-restauration montrait que les faibles salaires et les heures supplémentaires non rémunérées étaient cités en tête des raisons expliquant les difficultés de recrutement du secteur. Pour rendre ces métiers plus attractifs, les accords de branche ou d'entreprise sont des leviers intéressants, mais il est indispensable de mobiliser d'autres moyens. Il faut conclure. C'est pourquoi j'aimerais savoir ce que le Gouvernement pourrait mettre en oeuvre- pourquoi pas avec le concours des

Je voudrais, quant à moi, évoquer plus spécifiquement la question de l'apprentissage, pour lequel de nombreuses offres de formation et de contrats de travail en alternance ne sont pas pourvues. Dans ma région, nombreux sont les lycées professionnels et les entreprises qui cherchent sans succès de jeunes apprentis, notamment dans les filières traditionnelles de l'hôtellerie-restauration, de l'alimentation, de l'industrie, mais aussi dans certaines filières plus innovantes, comme le numérique.

Cette année encore, plus de 33 000 jeunes de ma région ont choisi l'apprentissage pour se former au métier de leur choix, dans l'un des 380 centres de formation. Mais c'est loin d'être suffisant ! Il faudrait 50 000 50 000 jeunes pour satisfaire les entreprises et remplir les formations. Comment améliorer cette situation ? Comment mieux communiquer auprès des jeunes pour revaloriser ces filières ? Car choisir l'apprentissage, c'est opter pour l'excellence, l'accès à une qualification reconnue et la perspective d'une insertion professionnelle rapide : près de 70 % des apprentis trouvent un emploi dans l'année qui suit l'obtention de leur diplôme.

avec les collectivités locales, les centres de formation et les entreprises afin d'attirer davantage de jeunes dans ces filières et formations d'avenir. La parole est Monsieur le sénateur, nous partageons cette conviction que l'apprentissage est l'une des grandes voies permettant de lutter contre le chômage massif des jeunes, véritable drame pour notre pays, pour les jeunes et pour leurs familles.

préfet. Pensez-vous que les préfets et les agents de l'État ont des consignes suffisamment pressantes et effectives pour s'atteler à cette dynamique économique, dont l'enjeu devrait être une priorité majeure ? La parole est à Mme la ministre.

des crédits de formation pour les demandeurs d'emploi en région Rhône-Alpes-une diminution de 65 % pour les bas niveaux de qualification -, nous ne sommes pas en mesure de signer ces formations, et c'est Pôle emploi qui prend le relais.

lui transmettre la passion d'un métier qu'il ne connaît pas et auquel il va s'identifier. Pour préparer la rentrée, le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer et moi-même avons écrit

propositions d'embauche sur dix sont en CDD ou en intérim. C'est probablement le problème majeur posé par nos règles d'assurance chômage, et notre priorité est de le régler. Bien évidemment, les partenaires sociaux ont toute liberté pour aller plus loin dans la réflexion. Peut-être feront-ils aussi des propositions sur ce sujet ?

En effet, 78 % des responsables de structures déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. Pourtant, il s'agit d'un secteur en pleine évolution. D'ici à 2030, le nombre d'emplois d'aide à domicile à pourvoir s'élèvera

est avancé comme la principale raison de ces freins, les contraintes de temps et d'organisation du travail, ainsi que la pénibilité, sont également largement mises en cause. C'est aussi le volume des personnes formées sur le territoire qui pose problème. Car aider les autres, c'est un métier, un métier, qui nécessite une vocation, certes, mais également une formation et un accompagnement. Madame la ministre, vous avez à coeur, je le sais, de porter des objectifs forts en matière de formation des salariés,

On est combien aujourd'hui ? » : c'est la question que se posent chaque jour des employés du secteur médico-social. Cette question cruciale dissimule à peine une surcharge de travail, des cadences intenables, des toilettes à réaliser à la hâte. La santé des soignants est en jeu tabagisme, maladies cardiovasculaires, stress, horaires décalés et invalidité font de ces métiers des professions à risques. Les syndicats des personnels estiment que 35 % des agents- infirmières aides-soignantes, aides médico-psychologiques, agents de service hospitaliers -, que ce soit dans le public ou dans le privé, ont le sentiment que l'effectif présent ne permet ni d'assurer la sécurité et la qualité des soins ni de respecter la dignité des patients.

ou plus. Au vu de ses besoins criants, madame la ministre, vous venez de vous prononcer sur des pistes. Mais j'aimerais vous entendre concrètement sur des améliorations à prendre en termes de reclassement, de déroulement de carrière, de rémunération et de protection sanitaire. Comment comptez-vous, madame la ministre, redonner leurs lettres de noblesse à ces métiers du soin ? La parole est

Luche. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, afin d'illustrer ce débat en parlant de ce que je connais le mieux, je vais prendre en exemple mon département de l'Aveyron.

Nous avons des atouts dans nos territoires ruraux : la sécurité, la proximité avec la nature, la qualité de vie, etc. Bien sûr, cela a été dit, la formation doit être améliorée, et la réforme de l'assurance chômage qui va être examinée par le Parlement sera déterminante pour favoriser le travail. Trouvons rapidement la solution à ce paradoxe : manque de travailleurs d'un côté, trop de demandeurs d'emploi de l'autre. Cela ne peut pas durer Par ailleurs, nous sommes plusieurs départements à vouloir attirer de nouvelles populations. Nous nous efforçons de nous faire connaître, de mettre en avant les qualités de nos territoires.

Pour nous, le développement économique et les nombreux emplois disponibles sont surtout liés à l'attractivité du territoire. Je sais toutefois que l'emploi dans nos territoires ruraux est nécessaire, mais pas suffisant. Pour cela, le maintien d'un service public de qualité est indispensable- je pense notamment à l'accès à la santé, à l'éducation et au très haut débit. Je reste persuadé qu'il faut investir aussi dans nos infrastructures routières, ferroviaires et numériques afin de favoriser la mobilité sur nos territoires. Les emplois non pourvus dans l'Aveyron pourraient enfin trouver preneur et, plutôt que de travailler dans les métropoles saturées, pourquoi ne pas créer un début d'exode urbain ? Madame la ministre, dans quelle mesure pouvez-vous prendre en compte l'aménagement du territoire afin d'aider nos chefs d'entreprise à recruter ? La parole est à Mme la ministre.

ruraux, des petites villes ou des villes moyennes était un véritable sujet, puisque beaucoup de ces habitants avaient le sentiment d'être loin des grandes métropoles où se concentrent l'emploi, l'activité,

parce que les entreprises, qui sont les mieux placées pour connaître leurs propres besoins, n'y occupent pas assez de place. Les entreprises trop éloignées de la formation, cela entraîne trois conséquences, que vous avez d'ailleurs évoquées : une inadéquation trop fréquente de la formation aux besoins réels, une méconnaissance totale par les jeunes de l'entreprise en général, de son fonctionnement et de son activité- vous avez dit qu'ils avaient une image datée des métiers et vous avez raison -, et enfin une méconnaissance de l'éventail des métiers et des opportunités de carrière. Or, dans la formation initiale, il existe un dispositif performant qui est l'apprentissage. Bon nombre des métiers en tension nécessitent un apprentissage. L'objectif de 500 000 places qui est régulièrement cité- je crois que vous l'avez fait vôtre -est toujours le même. J'ai entendu votre engagement ; néanmoins, nous stagnons depuis des années à 300 000 Avant de faire décoller l'apprentissage, encore ne faudrait-il pas l'entraver. Sur les 300 000 apprentis, 100 000 sont formés dans des centres de formation et des écoles dépendant des chambres consulaires. Or, loi de finances après loi de finances, le Gouvernement assèche véritablement ces chambres consulaires, poursuivant en cela la politique du précédent quinquennat. Pour 2018, la recette affectée est réduite de 100 millions d'euros. Le ministre de l'économie, Bruno Lemaire, a déclaré devant notre commission des affaires économiques qu'il ne faudrait pas que cette réduction ait un effet négatif sur les CFA et les écoles, et il l'a répété ce soir lors de de loi PACTE, mais il ne nous a pas dit comment. En l'état actuel, les CCI vont être contraintes de fermer des centres de formation, de se détourner de l'apprentissage au profit de la formation continue ou de la formation d'étudiants étrangers, plus lucratives. Ma question est simple : comment ferez-vous pour garantir que le nombre d'apprentis des chambres consulaires non seulement ne diminue pas, mais augmente de deux tiers comme il conviendrait pour atteindre nos objectifs ? La parole est à Mme la ministre. Madame la sénatrice, en ce qui concerne l'appareil de formation et notamment les centres de formation d'apprentis, nous avons complètement libéré, dans la loi Avenir professionnel,

une chambre consulaire, une profession, une entreprise pourra créer ou développer un CFA. Je peux vous dire que le nombre de projets en cours est très important. Par ailleurs, vous avez évoqué les organismes consulaires, qui assurent une grande partie de l'apprentissage aujourd'hui. La réforme prévue dans la loi Avenir professionnel va

de M. le Président de la République lors des Journées du patrimoine. Mes collègues l'ont déjà dit, l'expression « traverser la rue » a marqué- c'est évident -les esprits. Ces mots avaient douloureusement entaché la personne du président, comme si le chômage était une question de choix personnel et de volonté. La question des emplois non pourvus participe de cette idée que le travail est là, à portée de main de tout demandeur d'emploi et qu'il suffirait que ce dernier s'en saisisse. Or, mes chers collègues, vous le savez, si les offres d'emploi publiées n'aboutissent pas, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de candidats. L'étude de Pôle emploi parue en décembre 2017 et intitulée « Offres pourvues et abandon de recrutement » l'explique très bien : sur les 300 000 offres n'ayant pas trouvé preneur, près d'un tiers ont fait l'objet d'un retrait à la suite d'un changement de stratégie de l'entreprise et 50 000 offres faisaient l'objet de recrutement en cours. Nous avons effectivement les mêmes chiffres. Pour les offres restantes, pouvons-nous tenter de renverser la logique induite par ce débat en posant la question de l'attractivité de l'emploi proposé ? En effet, quelles sont les offres d'emplois qui ne trouvent pas preneur ? On a cité les contrats courts, les CDD de moins d'un mois, dont le nombre a explosé, les horaires décalés, les contrats dont la faible rémunération ne couvre pas les coûts induits ne couvre pas les coûts induits par ce travail- voiture, carburant, frais de garde, etc. Les « gilets jaunes » ont également confirmé que la mobilité était un enjeu fondamental, notamment en milieu rural. rural. Je le constate dans la Sarthe. En outre, l'expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » prouve que l'emploi est d'abord une question d'accompagnement social et permet de démythifier la rhétorique trop entendue des emplois non pourvus. Il est d'ailleurs très regrettable que l'exécutif n'ait pas étendu cette expérimentation à d'autres territoires dans le projet de loi de finances pour 2019. Ainsi, madame la ministre, vous avez affirmé précédemment vouloir envisager d'adapter le logiciel du marché du travail en termes d'attractivité des métiers, de mobilité et d'accompagnement. Pouvez-vous nous éclairer sur les moyens concrètement investis dans ces trois domaines, sans que cela pèse trop, bien évidemment, sur les collectivités locales, déjà fortement mises à contribution ? La parole est à Mme la ministre.

correspond à une conviction profonde, porte sur le tissu associatif très riche de notre pays, qui sait accompagner des chômeurs de longue durée, des anciens SDF, des personnes en situation de handicap. Ce sont les entreprises adaptées pour le handicap, ce sont les chantiers d'insertion et l'insertion par l'activité

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avec près de 6 millions de demandeurs d'emploi en France, on peut légitimement s'interroger sur les métiers qui demeurent en tension aujourd'hui. En effet, les difficultés de recrutement que rencontrent 23 % des entreprises durant le premier semestre 2018 mettent en lumière des phénomènes endémiques. Ainsi, 70 % des entreprises ayant eu du mal à recruter évoquent des problèmes de qualification évoquent aussi l'absence de candidatures. La part des embauches jugées difficiles s'accentue et s'élève à 44,4 % en 2018, tous secteurs confondus. Ces difficultés ont augmenté le plus dans les entreprises d'un à quatre salariés. salariés. Elles sont bien sûr liées à la pénurie de candidats, à l'inadéquation des profils, mais aussi aux conditions de travail. Pour les métiers de bouche par exemple, les projets de recrutement sont jugés difficiles à 74 % dans la boucherie, à 72,9 % chez les charcutiers-traiteurs, à 67 % en boulangerie-pâtisserie. Si l'on sait que ce déficit d'attractivité s'explique en partie par la priorité donnée à l'enseignement général au détriment des métiers de l'économie de proximité, où les opportunités sont pourtant plus nombreuses, on peut donc attendre de la part du Gouvernement des actions fortes visant à corriger ce phénomène. Alors que le besoin de main-d'oeuvre existe réellement dans les TPE artisanales notamment, comme dans le secteur du BTP, je vous demande, madame la ministre, de bien vouloir m'indiquer les dispositions qui sont prises pour accroître l'attractivité de ces métiers. La parole est

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 16 septembre dernier, un échange entre Emmanuel Macron et un jeune horticulteur en recherche d'emploi a relancé la question des emplois non pourvus. Dans un contexte de chômage élevé, l'existence d'emplois ne trouvant pas preneur est un paradoxe fréquemment dénoncé en France. Si le chiffre de 300 000 emplois non pourvus est souvent avancé, en réalité aucun indicateur ne permet aujourd'hui de mesurer l'ampleur réelle du phénomène ni d'en analyser les causes.

fait état d'une hausse inédite de 18,7 % du nombre de projets de recrutement, soit une augmentation de 370 000 par rapport à 2017. Près de 2 350 000 projets de recrutement étaient ainsi anticipés pour l'année 2018. Les plus fortes augmentations d'intentions d'embauche se situent dans la construction et l'industrie, avec des hausses respectives de 37 % et 27,4 %. Si ces chiffres sont plus qu'encourageants, cette même étude révèle malheureusement que les difficultés de recrutement perçues par les employeurs sont nettement en hausse. et des industries de l'hôtellerie, l'UMIH, entre 50 000 et 100 000 emplois n'ont pas été pourvus à l'été 2018. Cela explique probablement pourquoi ce début de reprise économique n'est pas encore perçu par les Français. 44,4 % des projets de recrutement sont jugés difficiles par les employeurs, contre 37,5 % l'an dernier. Selon les recruteurs, les candidatures inadéquates demeurent le principal motif de ces difficultés- soit l'employeur constate une pénurie de candidats, soit les profils ne lui conviennent pas. Se pose alors la question de l'employabilité de certains candidats et de l'attractivité de certains emplois, qui atteint même le recrutement des apprentis en CFA. Il est important d'encourager la reprise d'activité. L'emploi doit être plus rémunérateur et valorisant que les minima sociaux. Pouvez-vous, madame la ministre, me préciser aujourd'hui le plan d'action que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour anticiper le besoin de main-d'oeuvre pour 2019 ? Compte tenu des secteurs qui vont recruter, ne faut-il pas encourager les AFPA plutôt que de les fermer ? La parole est à Mme la ministre.

permettra aussi de montrer l'attractivité des métiers, y compris les métiers techniques et ceux de l'aide aux personnes. Il y a toutes sortes de métiers dans l'apprentissage, et chaque fois qu'on promeut l'apprentissage, on promeut le travail, on promeut la valeur du travail et on promeut l'attractivité des entreprises. La parole est à M. Yves Bouloux.

parmi les paradoxes français, le problème des emplois non pourvus n'est pas le moindre, alors que le taux de chômage est encore à plus de 9 %. Leur nombre pose une sérieuse question sur l'efficacité de notre politique de l'emploi et la vitalité de notre économie. Selon Pôle emploi, sur 300 000 offres d'emploi non pourvues en France, 97 000 ont été annulées, du fait de la disparition du besoin ou d'un manque de budget disponible dans les entreprises ; 53 000 n'ont pas abouti et sont encore en attente de recrutement, et 150 000 ont été abandonnées, faute de candidats. que j'ai exactement les mêmes chiffres que notre collègue Joël Guerriau. Les 150 000 abandons ne sont pas seulement le reflet d'un dysfonctionnement du marché du travail. Madame la ministre, quatre raisons peuvent expliquer ces abandons par les recruteurs.

Que comptez-vous faire pour les autres filières ? Deuxièmement, le manque d'attractivité des postes. Comment l'État pourrait-il concourir à l'attractivité de certains métiers et de certains secteurs et branches d'activité ? Troisièmement, l'inexpérience des recruteurs et leur méconnaissance du marché du travail. Prévoyez-vous la mise en place d'aides spécifiques aux employeurs les moins autonomes, PME et TPE en premier

J'ajouterai en outre trois autres questions. Comment adapter le contrôle des chômeurs à la réalité des emplois non pourvus ? Quelle réponse spécifique pouvons-nous apporter pour les départements et régions d'outre-mer ? Enfin, pensez-vous pouvoir améliorer la problématique des emplois non pourvus par des actions à l'échelle européenne, avec l'appui du réseau EURES ? La parole

Et pourtant, dans le même temps, la pénurie de compétences est devenue une des préoccupations majeures des entreprises. Plus d'un tiers d'entre elles ne parviennent pas à recruter les salariés dont elles ont besoin. Dans le cadre de la récente enquête « Besoins en main-d'oeuvre 2018 », Pôle emploi estime à 44,4 % la proportion de recrutements jugés difficiles par les entreprises en 2018, contre 37,5 % en 2017. 744 354 projets de recrutement sont considérés comme difficiles cette année. On estime par ailleurs que plus de 300 000 offres d'emploi restent non pourvues, faute de candidature. Cette situation est d'autant plus choquante qu'elle est incompréhensible. Certains feront porter la responsabilité sur les entreprises, en mettant en avant la dureté des conditions de travail dans certains métiers ou la faiblesse des salaires proposés. D'autres justifieront cette situation par l'inefficacité actuelle du dispositif de formation professionnelle. D'autres, enfin, considéreront que rien n'est fait pour inciter les demandeurs d'emploi à retrouver le chemin de l'entreprise et que les abus sont multiples. En réalité, l'ensemble de ces arguments sont sans doute à prendre en compte. Aucun secteur n'échappe au problème et il existe des pistes à creuser. La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle est une forme de réponse. Rappelons qu'elle consiste à identifier une compétence et à former une personne en vue d'une offre d'emploi disponible. Plus de 85 % des salariés entrant dans ce dispositif ont retrouvé un emploi. Sa généralisation pourrait être envisagée. Autre piste à explorer, l'incitation à la reprise d'emploi. Est-il, par exemple, acceptable qu'un salarié qui se voit offrir un CDI à l'issue de son CDD puisse le refuser et faire le choix de s'inscrire à Pôle emploi ? dit, il nous faut davantage miser réellement sur l'apprentissage, dont l'efficacité n'est plus à démontrer, mais qui peine toujours à s'imposer. On le voit, mes chers collègues, cette question difficile passe obligatoirement par un éventail de solutions. Il faut donc la traiter dans sa globalité en imaginant une chaîne de réponses multiples. Il est maintenant très urgent d'agir ! La parole est à Mme la ministre. Monsieur le sénateur, je partage tout à fait votre point de vue. Tous ceux qui pensent qu'il y a une baguette magique et une seule pour la lutte contre le chômage se trompent. vous qu'il y a un éventail de solutions. Il faut agir sur tous les leviers à la fois : l'offre, la demande, la formation, la mobilité, la motivation, la dignité du travail, les formes et conditions du travail. Bref, et, d'ailleurs, l'ensemble de vos questions le montrent, lutter contre le chômage de masse, c'est en même temps valoriser le travail, le retour au travail

de la construction sont les premiers concernés, mais il y a aussi la filière des services à la personne, le commerce, les TPE, les emplois saisonniers, en horaires décalés, et le travail le week-end. En décembre 2017, le conseil d'administration de Pôle emploi constatait que 150 000 à 200 000 offres n'étaient pas pourvues,

tandis que l'Allemagne compte 1,4 million d'apprentis et seulement 7 % de jeunes au chômage. Mon collègue Jean-Pierre Decool a fait état des difficultés de recrutement des apprentis dans certaines filières, notamment l'hôtellerie-restauration.

dans d'autres pays, comme en Finlande, l'orientation est pleinement intégrée dès l'école élémentaire, avec également, au collège, des visites dans les entreprises, des films sur les métiers et des entretiens individuels assurés par un enseignant spécifique. En ce qui concerne la formation, seulement ouvriers en font la demande à l'employeur, contre 50 % des cadres. La réalisation d'entretiens professionnels dans les TPE serait souhaitable. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel apporte des solutions pour les apprentis,

Actuellement, les CFA et les lycées professionnels sont gérés respectivement par les branches et l'éducation nationale, qui doivent travailler ensemble pour tenir compte de la spécificité de l'emploi des territoires et faire de l'apprentissage une voie d'excellence. Il est nécessaire d'associer Pôle emploi, la région, les partenaires sociaux et les entreprises pour réorganiser la formation, en particulier en tenant compte des compétences recherchées dans les bassins d'emploi. Le Gouvernement a misé sur la formation professionnelle, avec un financement de 15 milliards d'euros entre 2018 2018 et 2022 pour rehausser le niveau de compétences des plus éloignés de l'emploi. L'aide à la mobilité, notamment dans le milieu rural, est essentielle. Il faut une différence de salaire suffisamment incitative, coût de mobilité compris, entre les personnes qui travaillent et celles qui restent inactives. Le réseau emplois compétences pourrait tenir le rôle de plateforme de coordination, chargée de centraliser, de traiter les données locales et d'anticiper les besoins par le déploiement de formations centrées sur les compétences recherchées dans les bassins d'emploi. Pour conclure, la lutte contre le chômage passe par la formation initiale et continue, notamment par une voie d'apprentissage, mais aussi par une coopération étroite avec les entreprises, les plus à même d'identifier les salariés dont elles ont besoin. Les personnes handicapées pourront, avec le doublement des entreprises adaptées, trouver aussi une solution. Redonner un sens et une valeur au travail, faire de l'apprentissage une voie d'excellence, favoriser les mobilités internes et géographiques, ainsi que les formations en entreprise : tels sont les principaux axes d'action que nous proposons pour apporter

La séance est levée.